règlement. Les projets de loi de financement de la sécurité sociale passent, et le droit parlementaire continue de décroître. Déjà, l'an dernier, notre groupe avait dénoncé le sort réservé aux amendements déposés par les différents groupes sur le PLFSS 2020. Pour rappel, 320 amendements avaient été déclarés irrecevables, dont 54 déposés par notre groupe. Cette année, 370 amendements ont été rejetés sur les 1 062 déposés, dont 33 des 97 de notre groupe. Si le durcissement des conditions de recevabilité des amendements a également été constaté à l'Assemblée nationale, nous souhaiterions que le droit d'amendement, qui est un principe à valeur constitutionnelle, soit respecté.

votre appréciation des contenus de nos amendements. Notre impression est que le durcissement des conditions de recevabilité des amendements revient à porter une atteinte accrue au droit d'expression des groupes parlementaires, singulièrement des groupes minoritaires d'opposition. Désormais, si nos amendements comprennent des mesures financières, et malgré la présence d'un gage financier, ils sont retoqués au titre de l'article 40 de la Constitution. Je donnerai deux exemples. Nous avions déposé un amendement

Pourtant, si le délai légal est prolongé, le nombre d'avortements risque mécaniquement d'augmenter, avec des conséquences financières en termes de prise en charge pour la sécurité sociale. Autre exemple : nous avions déposé un amendement tendant à créer un programme public de production et de distribution du médicament. Il a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40, alors qu'il visait à augmenter la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques. J'appelle solennellement les groupes politiques à prendre conscience de la réduction en cours du droit d'opposition et du droit parlementaire d'amendement. Défendre les droits du Parlement, c'est commencer par garantir le droit d'amendement,

de ne pas compenser les exonérations de cotisations sociales, donnant un prolongement aux conclusions du rapport dit « Charpy-Dubertret » sur la rénovation des relations financières entre l'État et la sécurité sociale. sociale. Si l'État avait tenu ses engagements et respecté la loi Veil et l'autonomie budgétaire de la sécurité sociale, le budget n'aurait pas été amputé de 4,3 milliards d'euros.

Faire participer ces organismes à l'effort financier national inhérent à la gestion de la pandémie nous semble donc une bonne mesure. Néanmoins, il convient d'opérer une distinction entre assurances privées et mutuelles, ces dernières étant, je vous le rappelle, des organismes à but non lucratif.

Il ne nous semble pas juste de leur imposer cette nouvelle fiscalité pour 2020 et 2021, et nous n'avons pas fait le même choix qu'Alain Milon, qui propose de différencier les taux.

Le rapporteur général de l'Assemblée nationale avait rétorqué à mon collègue Pierre Dharréville, qui défendait un amendement similaire, que cette proposition était contradictoire avec notre volonté de ne pas assécher les recettes de la sécurité sociale.

le code de la sécurité sociale ou le code rural et de la pêche maritime. Il s'agit d'instaurer une différenciation dans la contribution exceptionnelle demandée en 2020 aux organismes complémentaires, selon qu'il s'agisse de mutuelles, sans but lucratif, ou de compagnies d'assurances privées, à but lucratif. Les compagnies d'assurances privées, qui couvrent d'autres marchés que celui des complémentaires santé, ont enregistré des surplus de cotisations importants

Je n'ai rien contre les mutualistes, bien au contraire- j'en suis ! -, mais je considère que tout le monde, en l'espèce, est à la même enseigne : les charges

l'avis du Gouvernement ? il ne s'agit pas de dire que les organismes mutualistes ou d'assurance complémentaire ont souhaité réaliser des économies à l'occasion de la crise, nous faisons simplement cette constatation -à 2,2 milliards d'euros, en tenant compte d'un phénomène de rattrapage des soins sur la dernière partie de l'année.

des secteurs économiques qui, eux, n'ont absolument aucun rapport avec la solidarité et qui ont engrangé des profits supplémentaires considérables.

vise à instituer un abattement de 50 % sur la contribution exceptionnelle des complémentaires de santé pour les cotisations qui sont versées par les entreprises du secteur de la culture. Vous savez à quel point les entreprises de ce secteur connaissent depuis le mois de mars dernier un arrêt quasi intégral de leur activité. Si plusieurs plans d'aide ont été engagés en faveur de ce secteur, les conséquences de cette crise sanitaire et économique sont telles que toute l'architecture de cet accompagnement social est aujourd'hui ébranlée par des cotisations sociales en baisse et des prestations de prévoyance qui menacent d'exploser.

diminuer la contribution des OCAM sur les sommes versées par des entreprises relevant des branches professionnelles de la culture. J'avoue ne pas trop comprendre ce que vient faire cette distinction en faveur des professionnels de la culture ... Il s'agit des OCAM

aux coûts suscités par la gestion de l'épidémie de covid-19 ne puisse être répercutée sur les régimes collectifs complémentaires pilotés par les branches professionnelles et hébergés par des organismes assureurs. Ces organismes doivent, par conséquent, financer cette contribution sur leurs fonds propres.

Alors que la pandémie du covid-19 a contraint les petits commerces à baisser les rideaux, les géants technologiques ne se sont jamais aussi bien portés. Notre collègue Éric Bocquet a d'ailleurs interpellé le Gouvernement, la semaine dernière, sur la question des rentes d'Amazon, qui ont augmenté de 26 % au premier trimestre 2020. Il a appelé à taxer, enfin, les bénéfices des géants du numérique

les librairies indépendantes. Cet amendement tend à s'inscrire dans la continuité de la taxe Gafam adoptée en 2020 par le Parlement et dont le recouvrement a été, je le rappelle, suspendu par le Gouvernement, pour, disait-il, « donner une chance aux négociations internationales » internationales » ... Les négociations ayant échoué, nous ne pouvons en rester là. Nous proposons de mettre à contribution les plateformes de qui ont profité des périodes de confinement pour réaliser des bénéfices exceptionnels. Il s'agirait pour nous d'une contribution ponctuelle pour cette année 2020, au taux de 0,5 %, pour financer les dépenses de santé liées à la pandémie du covid-19. Quel

mise en place par la France pour l'année 2020. Le montant devrait être- je parle au conditionnel, ne maîtrisant pas totalement la base d'imposition à ce stade -, autour de 350 millions d'euros, comme l'année précédente. Ainsi, la France, comme nous nous y étions engagés lors du PLF 2019, à la fin de l'année 2018, a créé une taxe sur les Gafam à hauteur de 350 millions d'euros, qu'elle a perçue en 2019 et qu'elle va percevoir en 2020, tout en continuant à porter ce sujet au sein de l'OCDE, avec la conviction toujours renouvelée que c'est au niveau international que nous aurons les meilleures réponses- les plus efficaces,

une distorsion de concurrence entre le commerce de proximité et ces plateformes, qui, elles, peuvent continuer d'alimenter les consommateurs français en produits non essentiels. Allons-nous continuer à les regarder

En effet, si la réforme permet à un assuré de bénéficier d'un équipement sans reste à charge, celui-ci n'en demeure pas moins contraint de devoir avancer les frais pour son acquisition, selon les conditions particulières d'accès au tiers payant intégral fixées par sa complémentaire de santé. près de 27 % des patients en optique et 57 % en audiologie n'ont pas accès au tiers payant intégral. Pour les Français les plus fragiles, cette avance de frais peut constituer un motif de renoncement aux soins, contre lequel le 100 % Santé doit justement permettre de lutter. certains organismes de complémentaire santé font de l'accès au tiers payant intégral un enjeu commercial et prudentiel, de nombreux bénéficiaires d'équipements inclus dans le 100 % Santé risquent de ne pas pouvoir en bénéficier. En effet, dans le cadre du contrat solidaire et responsable, les organismes complémentaires ont pour seule obligation d'assurer le tiers payant sur le ticket modérateur. C'est pourquoi le présent amendement vise à conditionner les avantages fiscaux accordés aux complémentaires de santé à la pratique du tiers payant intégral. Il tend également à prévoir des sanctions en cas de non-respect de cette obligation, tant pour les complémentaires que pour les professionnels de santé. De telles dispositions sont nécessaires pour assurer le plein succès de la lutte contre le renoncement aux soins pour des raisons financières ; c'était un engagement fort du Président de la République.

en adaptant la correction de leurs patients après la réalisation d'un examen de la réfraction. Cette prestation participe très largement à l'amélioration de l'accès aux soins visuels, puisqu'elle donne lieu à un remboursement à 100 dans le cadre du panier de soins. Cependant, cette même prestation n'est plus remboursée par les organismes complémentaires lorsqu'elle donne lieu à la délivrance d'un équipement en dehors du 100 % Santé,

n° 65 rectifié. Cet amendement vise à encadrer la pratique du remboursement différencié dans le cadre du contrat solidaire et responsable. Cette pratique permet aux complémentaires de moins bien rembourser leurs assurés qui ne se rendraient pas chez un professionnel de santé affilié à leur réseau de soins, y compris lorsque celui-ci est leur professionnel de santé habituel. Le niveau de remboursement des assurés peut varier, par conséquent, du simple au double chez certaines complémentaires de santé. Par ailleurs, cette pratique va à l'encontre des objectifs fixés par la loi. Cet amendement a donc pour objet d'apporter des conditions aux avantages fiscaux accordés aux complémentaires de santé, en limitant le niveau possible de différenciation des remboursements dans et hors réseau de soins.

Il s'agit ici de majorer de 7 points la taxe de solidarité additionnelle, la TSA, pour les OCAM qui proposent des différenciations,

en fonction du recours, ou non, à un réseau de soins ne nous paraît pas souhaitable, les réseaux de soins autorisant régulièrement des économies d'échelle qui nous paraissent intéressantes. L'adoption de l'amendement n reviendrait à mettre en cause l'équilibre de négociation trouvé avec les OCAM dans le cadre de la mise en oeuvre du reste à charge zéro. Nous ne souhaitons pas contrarier, si vous me passez l'expression, cet équilibre de négociation.

Décidément, 2020 est une année très particulière ! La survenue de la pandémie a bousculé le quotidien des Françaises et des Français. Des expressions nouvelles sont apparues : la « première ligne » et la « deuxième ligne », expressions qui filent la métaphore guerrière du Président de la République, par opposition à celles et ceux qui se retranchaient à leur domicile pour contenir la propagation du virus. Certains métiers sont soudainement apparus comme essentiels à celui qui n'avait d'yeux que pour « les premiers de cordée En première ligne se trouvent les soignantes et les soignants des hôpitaux, applaudis, mais aussi les employés de l'aide à domicile, indispensables pour pallier la perte d'autonomie de ceux qui vieillissent chez eux, ou encore les auxiliaires du quotidien des personnes en situation de handicap. L'attribution d'une prime covid pour rétribuer ses personnels a pris du temps. La doctrine, le « quoi qu'il en coûte », est plus simple à formuler qu'à appliquer. Un accord conclu en août dernier entre l'État et les départements de France a abouti à une prise en charge de la prime covid pour les personnels de l'aide à domicile. de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, en contrepartie du même effort consenti par les conseils départementaux. Les socialistes soutiendront ce financement de la prime covid, par égard pour les salariés mobilisés, mais nous formulons des remarques. Son financement repose sur les 50 millions d'euros qui avaient été ouverts afin d'esquisser une réforme du financement de l'aide à domicile et des services d'accompagnement et d'aide de cette expérimentation n'est pas un bon signal au regard du chantier de l'autonomie qui est devant nous. Nous avions proposé un amendement pour ne pas y renoncer, mais il a été jugé irrecevable. Pour nous, cette rallonge de 80 millions d'euros est clairement insuffisante au regard de l'ensemble des surcoûts rencontrés par les services d'aide à domicile, difficilement équipés en masques par les dotations des ARS. Les associations elles-mêmes ont engagé des frais imprévus pour acheter des gants, des masques et des surblouses, et ainsi protéger le personnel, en même temps que leurs recettes diminuaient. Les représentants des SAAD estiment à 265 millions d'euros le besoin de financement nécessaire pour équilibrer les dépenses engagées durant la crise. Nous sommes loin du compte

sur le versement de la prime aux personnels dont vient de parler ma collègue Michèle Meunier. Nous n'avons pas attendu, malgré les difficultés que nous pouvons éprouver dans certains départements, et bien que l'État nous soit encore très fortement redevable, au regard de toutes les allocations individuelles que nous versons et qui sont loin d'être compensées. Ce retard est certes très ancien, mais aucun gouvernement- celui-ci non plus -ne l'a rattrapé. Le Gouvernement a suivi, en prévoyant cette aide qui est insuffisante. Cependant, j'irai plus loin. Ce n'est pas une aide complémentaire que nous sollicitons, mais tout simplement

des caisses de retraite et des mutuelles. Or, si seule la prise en compte des heures financées par les départements sert de critère éligible pour les modalités de calcul du montant de la prime, de fortes injustices seraient constatées pour des personnels ayant travaillé une majeure partie de leur temps pour des plans d'aide « caisse de retraite » ou « mutuelle »- ils ne toucheraient cette prime 318 rectifié vise à rendre éligible à la prime covid à taux plein l'ensemble des personnels SAAD mobilisés durant la crise sanitaire.

rapport ne me paraît pas nécessaire, d'abord parce que la CNSA, dont les missions sont clarifiées par le présent texte, pourra exercer ce rôle d'évaluation, et, ensuite, parce que le Parlement a la possibilité d'évaluer lui-même de tels dispositifs-

Les publics fragiles accompagnés, souvent âgés, handicapés ou dépendants, sont particulièrement vulnérables à la covid-19, et ces services ont dû faire preuve d'une capacité d'adaptation inédite, tandis que les agents sont souvent précaires et difficiles à recruter. Les départements sont en première ligne dans la prise en charge de la dépendance et de la perte d'autonomie. Or ils sont aujourd'hui doublement pénalisés par l'explosion des dépenses, d'une part, et le manque de soutien financier des crédits d'État, d'autre part. L'exonération « aide à domicile » vise un double objectif : assurer la prise en charge des personnes fragiles ; soutenir et dynamiser l'emploi dans un secteur d'activité en pleine explosion. L'application du dispositif peut entraîner jusqu'à 27 % de réduction de charges patronales pour un employeur des professionnels concernés, et les départements, qui devraient être parmi les premiers à bénéficier de cette exonération, s'en trouvent aujourd'hui exclus pour diverses raisons.

n'est pas définie en droit de la sécurité sociale, et c'est pour cette raison que les Urssaf ont rejeté les demandes d'exonération d'autres catégories d'établissements, comme les foyers d'accueil médicalisé, les FAM, ou les foyers de vie, au motif qu'il ne s'agirait pas strictement d'un domicile privatif. De nombreux établissements éligibles non médicalisés, financés non pas par la sécurité sociale, mais par les départements, se trouvent ainsi exclus du champ d'application L'objet de cet amendement est donc de clarifier les critères d'éligibilité des établissements susceptibles de bénéficier d'exonération en supprimant la notion trop floue, pour les Urssaf, de domicile privatif, pour se concentrer sur la nature des tâches effectuées.

à domicile. Ce mécanisme, introduit par la LFSS pour 2019, est une exonération supplémentaire de cotisations pour les structures intervenant dans cette aide à domicile. Elle est dégressive, entre 1,2 SMIC et 1,6 SMIC, et limitée aux structures privées. L'objet de l'amendement dénonce les disparités entre le secteur public et le secteur privé, ce à quoi l'on peut souscrire, mais son dispositif se contente de limiter cette exonération aux structures à but lucratif, ce qui semble, pour moi, quelque peu en contradiction avec le but visé. En toute hypothèse, l'impact sur l'emploi de ce mécanisme et l'impact financier de cet amendement mériteraient d'être évalués, avant d'envisager une modification du périmètre. Nous sollicitons donc l'avis du Gouvernement sur ce point.

Les CCAS et CIAS bénéficient d'une exonération des cotisations de sécurité sociale, hors AT-MP, soit un taux d'exonération de 28,7 % applicable sans plafond de rémunération et sans dégressivité. votre demande est donc déjà satisfaite s'agissant des CCAS et des CIAS. En revanche, comme le disait M. le rapporteur général, introduire une distinction, au sein des établissements de droit privé, entre les établissements à but lucratif et ceux à but non lucratif risquerait de créer une rupture de l'égalité devant l'impôt. Je n'y suis donc pas favorable.

que les activités financées par des organismes de sécurité sociale sont exclues du dispositif d'exonération. L'objet de cet amendement est donc de clarifier les critères d'éligibilité des établissements pouvant bénéficier de l'exonération, en supprimant la notion, trop floue pour les Urssaf, de domicile privatif, pour se concentrer sur la nature des tâches effectuées.

de charges par les établissements à but non lucratif a pour objet d'assurer la bonne application de la règle de droit, il ne doit pas avoir pour effet d'empêcher systématiquement son application. Si un employeur à but non lucratif est éligible, que les activités réalisées sont éligibles et que l'ensemble des bénéficiaires est également éligible, il n'est ni opportun ni nécessaire de justifier avec une précision abusive les heures de travail de ces agents. L'objet de cet amendement est donc de dispenser les établissements à but non lucratif de l'application de règles de preuve inutiles adaptées pour le secteur lucratif, dont la production confine à l'impossible.

. Je rejoins ce que vient de dire M. Bonne, donc je vais être beaucoup plus courte. Si un employeur à but non lucratif est éligible, que les activités réalisées sont éligibles et que l'ensemble des bénéficiaires est éligible, il n'est ni opportun ni nécessaire de justifier avec une précision abusive les heures de travail de ces agents. L'objet de cet amendement est donc de dispenser les établissements à but non lucratif de l'application de règles de preuve inutiles, adaptées par le secteur lucratif, dont la production confine à l'impossible. Quel est l'avis de la commission

C'est bien l'apport d'un justificatif qui permet de déterminer si la personne auprès de laquelle intervient l'aide à domicile est fragile. L'absence de justificatif, à terme, conduirait à une application automatique à tout le monde de l'exonération, qui est normalement réservée aux personnes dépendantes.

l'on peut changer aussi facilement la donne. Pour autant, j'y insiste, ne partons pas du postulat que toutes les personnes que vous avez évoquées sont les bénéficiaires uniques de ces prestations.

La situation en mars dernier a en effet justifié de relever ces plafonds à un niveau jamais égalé. Les reports de cotisations accordés aux employeurs et aux indépendants culminaient à 16,6 milliards d'euros pour les employeurs à la fin juin, et à 18,3 milliards d'euros pour les indépendants à la fin août. Autant de recettes en moins pour l'Acoss, alors que, dans le même temps, les dépenses de l'assurance maladie grimpaient en flèche. La situation était si inédite que la limite dans laquelle les régimes obligatoires de base pouvaient recourir à des ressources non permanentes pour couvrir leurs besoins en trésorerie aurait été dépassée dès le début du mois d'avril si rien n'avait été fait. Ces plafonds ont donc été révisés en mars, puis en mai, dans des proportions jamais atteintes : 95 milliards d'euros, soit +144 % par rapport au plafond que nous avions fixé dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. La loi organique prévoit qu'il puisse être dérogé au montant fixé en loi de financement par décret, mais elle prévoit également, premièrement, que la ratification de ce décret soit demandée au Parlement dans le plus prochain PLFSS,

ailleurs, les montants inédits dont nous parlons auraient justifié de nous présenter un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale en cours d'année. La ratification de ces décrets en aurait été, en partie, l'objet.

que le Gouvernement daigne se montrer respectueux de ses obligations constitutionnelles. C'est pourquoi nous n'accepterons pas de ratifier ce dépassement en votant cet article 5.

est passé de 150 millions d'euros- nous n'étions déjà pas tout à fait d'accord -à 4,8 milliards d'euros, du fait de la nécessité de procéder à des achats massifs de divers matériels médicaux pour répondre à la crise sanitaire. Cela confirme Cela confirme la pertinence de l'analyse du Sénat, qui s'était opposé à ce transfert l'année dernière. Il convient,, que la sécurité sociale soit compensée à due concurrence des coûts extraordinaires

Nous considérons que le fait d'intégrer Santé publique France dans le périmètre de la sécurité sociale se justifie pleinement par la nature même des activités et des services attendus de cet organisme. mis en place ce nouveau « périmétrage », si j'ose dire, il a été prévu une compensation par une fraction de TVA. Je le concède bien volontiers, cette mise en place s'est faite hors épidémie. Vous le dites vous-même, la première année se caractérise par la nécessité de faire face à l'épidémie, avec des dépenses qui sont, certes, importantes, mais qui, nous le souhaitons tous, sont conjoncturelles.

de la sécurité sociale, dans les conditions qui avaient été pensées hors crise, considérant que ce que nous connaissons aujourd'hui est tout à fait conjoncturel.

qui s'est déroulé sur plusieurs années et qui a amené l'État à transférer progressivement le financement des différentes agences sanitaires vers l'assurance maladie-

Par ailleurs, concernant plus spécifiquement l'Agence nationale de santé publique, j'observe qu'elle remplit nombre de missions qui sont non pas du ressort de la sécurité sociale, de l'assurance maladie, mais de strictes prérogatives de l'État.

je crois que ce n'est pas la réponse la plus satisfaisante. Pour nous, la réponse satisfaisante, c'est de dire que l'Agence nationale de santé publique relève bien du domaine de l'État. Par ailleurs, la crise que nous vivons actuellement doit nous amener à revisiter l'architecture générale, celle de l'État, de ses agences, des lieux où s'exercent les compétences en matière sanitaire, et de leur articulation. La parole

Il était donc nécessaire de simplifier son application ; on permet ainsi aux employeurs d'en bénéficier plus facilement. Le dispositif mis en place dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prévoyait que les indemnités d'activité partielle ne soient assujetties à la CSG et à la CRDS applicable aux revenus de remplacement. L'article que nous examinons, issu des débats de l'Assemblée nationale, pérennise l'activité du régime social des indemnités d'activité partielle au-delà du 31 décembre 2020, la mesure de validation du trimestre de base au titre de l'activité partielle. Il était essentiel de permettre de sécuriser les droits sociaux des assurés qui bénéficient de ce dispositif. C'est pourquoi nous nous réjouissons de l'introduction de ces nouvelles dispositions,

Un certain nombre de dispositifs de report, puis de réduction des cotisations sociales ont été mis en place pour aider les entreprises et les salariés de ces secteurs. Alors que de nouvelles mesures de restriction de l'activité ont été mises en oeuvre afin d'endiguer la circulation du virus et de protéger les Français les plus exposés, il est urgent de venir compléter

en prévoyant un dispositif complémentaire d'exonération au bénéfice des entreprises du secteur dit « S1 », c'est-à-dire de celles qui ont fermé totalement ou qui sont situées dans des zones de couvre-feu et qui ont subi une baisse d'activité significative. Je pense enfin au dispositif de réduction forfaitaire mis en place pour les travailleurs indépendants. Ces dispositions sont plus que nécessaires au regard des difficultés que rencontrent un certain nombre d'entreprises de ces secteurs ; elles nous paraissent évidentes et essentielles : c'est pourquoi nous les soutiendrons.

la condition de baisse d'activité est ramenée de 80 % à 50 % pour l'ensemble des entreprises dépendant des secteurs les plus affectés, dits « liste S1 ».

Pris dans sa globalité, le dispositif pourra représenter jusqu'à trois mois d'exonération, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, dont un mois au titre du couvre-feu qui a été mis en place au mois d'octobre. Les restrictions, ainsi que les conditions de baisse d'activité, seront appréciées d'octobre à décembre, et les cotisations exonérées seront également celles qui sont exigibles d'octobre à décembre, c'est-à-dire celles qui portent, chaque mois,

Cette solution, qui avait déjà été retenue au moment du premier confinement, est en pratique plus favorable ; elle permet d'exonérer les entreprises de cotisations en fonction du moment où elles sont effectivement dues par les employeurs. Dans le détail, le dispositif bénéficiera en premier lieu aux entreprises de moins de 250 salariés des secteurs les plus affectés par les restrictions- l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, la culture, le sport, l'événementiel et le transport aérien -, puisque ces secteurs ont été directement touchés par le couvre-feu ou le confinement- nous avons pris l'habitude de les

Enfin, le dispositif mis en place au titre du confinement sera applicable dans l'ensemble des collectivités d'outre-mer, même si le confinement n'y est pas localement applicable : je le dis en réponse à l'amendement n° 729 rectifié de Mme Jasmin, qui se voit ainsi satisfait. Comme au printemps dernier, les entreprises concernées bénéficieront d'une exonération totale des cotisations sociales patronales, hors retraite complémentaire, exigibles le mois où les conditions d'éligibilité sont remplies. Elles bénéficieront aussi d'une aide égale

visant à appliquer ce système d'exonérations aux entreprises de plus de 250 salariés recevront un avis défavorable du Gouvernement, car d'autres dispositifs existent pour les entreprises plus grandes que les TPE et les PME.

vous l'avez rappelé -exclus de ce dispositif. Non, je parle ici de tout l'écosystème, si fragile, des clubs de volley-ball, de hockey sur glace, de basket-ball, de handball, de rugby, ou de football qui tentent de survivre. Je parle des sports professionnels masculins, mais aussi et surtout des sports professionnels féminins, dont le modèle économique est fondé presque uniquement, soit sur le soutien des collectivités, soit sur les recettes de billetterie et les contrats de partenariat avec les espaces de convivialité.

dans le cas où les compétitions sportives professionnelles se déroulent dans des enceintes sportives dont la jauge d'accueil aura été limitée, par le Gouvernement, à mille personnes ou moins, ou encore à huis clos, ce qui est le cas aujourd'hui.

L'objet de cet amendement est donc, d'une part, de baisser à 70 % le seuil de perte de chiffre d'affaires à partir duquel une entreprise dépendante peut bénéficier de l'exonération totale de cotisations, et, d'autre part, de créer un dispositif d'exonération partielle par palier en fonction de la perte de chiffre d'affaires de ces entreprises.

plus largement en compte les difficultés rencontrées par ces entreprises, le seuil de 80 % étant trop élevé pour intégrer

que j'ai cités peuvent être en difficulté et que les clubs de moyenne importance, qui sont absolument indispensables à la vie des territoires,

du Gouvernement ?

En l'état de la rédaction du sous-amendement, l'absence complète de référence à l'effectif des sociétés qui exercent dans le domaine sportif ouvre le champ

qui ouvre 115 millions d'euros de crédits pour accompagner les structures sportives qui perdent des recettes de guichet du fait de la limitation des jauges. Nous avons pour objectif, non pas de soutenir les plus grandes sociétés sportives que vous avez évoquées, mais bien de nous focaliser sur l'ensemble des clubs que l'on qualifie parfois de « semi-professionnels » : on sait combien les recettes de guichet sont importantes dans leur chiffre d'affaires et leur revenu global. Enfin, il y a une troisième raison, que j'ai déjà évoquée

: ce sera introduit dans la doctrine et dans les instructions ; les employeurs qui exercent dans le domaine sportif et qui répondent à ce que vous avez décrit dans votre présentation de l'amendement, donc à vos objectifs, seront accompagnés. Nous tiendrons compte de la réduction de la jauge et de la réduction capacitaire

en l'espèce et sans commenter la philosophie ni l'orientation générale de votre propos, votre argument tiendrait si le Gouvernement n'avait pas déjà pris l'engagement de compenser, auprès de la sécurité sociale, les exonérations de l'article 6 , comme celles du PLFR 3 : celui-ci avait permis de voter simultanément

Alors que la tenue de salons nécessite un cycle de production de six à huit mois minimum, l'absence totale de visibilité et de prévisibilité quant à la réalisation effective de ce type d'événements empêche d'envisager tout redémarrage avant le mois de septembre 2021. Afin de soutenir la petite dizaine d'entreprises de taille intermédiaire de cette filière, qui constituent des moteurs essentiels pour tous les maillons de la chaîne de valeur, il apparaît nécessaire de relever le seuil permettant de bénéficier de ces exonérations, de 250 à 500 salariés. Les établissements recevant du public de type T ayant fait l'objet d'une fermeture administrative jusqu'à la fin du mois d'août et l'organisation d'événements ayant par la suite fait l'objet de restrictions quant au nombre de personnes pouvant être accueillies simultanément, il convient d'accorder le bénéfice de cette exonération, dès le mois de juin 2020, non seulement aux activités ayant fait l'objet d'une fermeture administrative, mais aussi à celles qui n'ont fait l'objet que d'une limitation administrative du nombre de leurs participants. Aussi, l'objet du présent amendement est d'accorder le bénéfice de l'exonération de charges sociales aux employeurs du secteur de l'événementiel de moins de 500 salariés, dont l'activité a fait l'objet d'une interdiction administrative d'exercer ou lorsqu'un seuil de personnes rassemblées simultanément a été fixé par l'autorité administrative, et ce dès le 1 juin 2020. Quel est l'avis de la commission

l'avis de la commission ? Le dispositif de l'article 6 est ouvert, d'une part, aux entreprises de moins de 250 salariés, et, d'autre part, aux travailleurs indépendants. Cela

rassurer les chefs d'entreprise qui considéreraient ne pas pouvoir honorer cette dette dans les délais impartis. En outre, nous proposons dans les dispositions ajoutées dans

J'étais ce matin à Nancy dans l'un des centres d'appels téléphoniques nationaux qui accueillent l'ensemble des demandes des entreprises de métropole et d'outre-mer.

le dispositif du fonds de solidarité aux entreprises n'existait pas : monté en dix jours, il a traité un 1,7 million de demandes. Les dispositifs de chômage partiel ont été totalement modifiés et les salariés ont été payés à chaque fois.

Mme Florence Lassarade. Cet amendement vise à apporter un soutien à la filière de la restauration aérienne qui souffre drastiquement à la fois de la baisse massive du trafic aérien et du nombre de passagers et de la réduction d'offres à bord par les compagnies aériennes. Sa survie est désormais en jeu, avec des milliers d'emplois à la clé. La majeure partie du chiffre d'affaires des opérateurs de la filière se fait sur des vols long-courriers qui sont très touchés par les différentes mesures prises par les États pour limiter l'accès à leur territoire, Les reports de charges obtenus au printemps et les prêts garantis par l'État (PGE) souscrits vont devoir commencer à être remboursés, alors même que la situation économique des entreprises est encore plus fragile plus fragile après une période de graves difficultés, sans perspective de reprise dans les mois à venir. L'Association internationale du transport aérien (IATA) ne prévoit pas de reprise normale du trafic équivalente à celle qui prévalait avant la pandémie de la covid-19 avant 2024. Un appui doit être mis en place de manière urgente pour permettre aux entreprises de restauration aérienne, qui sont fortement affectées par la crise, de préserver l'emploi coûte que coûte, notamment dans les différents aéroports parisiens et de province très durement touchés. Ce soutien à l'emploi et à la filière doit se matérialiser par une exonération complète des charges sociales, patronales et salariales, pour l'année 2021.

Le ministre nous l'a rappelé : l'Assemblée nationale examine le quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2020. Le budget de la sécurité sociale devait-il à ce point se passer de l'avis du Parlement durant toute cette année ?

des prélèvements sociaux sur le capital affecté au Fonds de solidarité vieillesse (FSV). Les soldes du régime général et du FSV pour 2020 sont ainsi dégradés de 2,4 milliards d'euros par rapport au texte adopté en première lecture à l'Assemblée nationale.

Vous avez refusé, prétextant qu'il n'y avait pas besoin d'un tel débat et que le PLFSS 2020 suffirait. Pourtant, le Sénat discute à présent d'un amendement de près d'un milliard d'euros

Nous nous apprêtons à voter un Ondam 2020 révisé à 218,9 milliards d'euros. J'insiste sur le caractère assez exceptionnel de cette discussion : nous en sommes déjà à la troisième proposition de révision de la part du Gouvernement.

Ce relèvement de 10,1 milliards d'euros tirait déjà les conséquences de surcoûts bruts liés à l'épidémie de covid-19, estimés alors à 15,1 milliards d'euros. Compte tenu de la dégradation de la crise sanitaire cet automne, le Gouvernement a relevé ce montant de 2,4 milliards d'euros à l'Assemblée nationale, et il nous propose à présent une troisième révision,

Après la parution du décret du 3 juillet 2018 portant dispositions applicables aux étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie, il est apparu, en septembre 2020, que les moyens budgétaires nécessaires n'avaient pas été mis en place à l'échelle des hôpitaux ni, de toute évidence, à une échelle supérieure, régionale ou nationale. Il en résulte des aménagements organisationnels pour supprimer purement et simplement le principe de supervision de ces docteurs juniors.

37 millions d'euros sont d'ores et déjà prévus dans l'Ondam 2020 pour la revalorisation des étudiants de deuxième et troisième cycles des études médicales, chirurgicales et odontologiques. En 2021, 154 millions d'euros supplémentaires seront consacrés aux revalorisations salariales des étudiants en médecine dans le cadre des engagements pris lors des accords de Ségur. Ces crédits vont permettre de financer la revalorisation des étudiants de deuxième cycle des études médicales, dont les émoluments ont été doublés en première année dès le 1 septembre, et celle des étudiants de troisième cycle,

de revenir devant le Parlement avant le mois de novembre pour corriger en tant que de besoin la loi de financement de la sécurité sociale ? La parole est à Mme Corinne

que le Gouvernement réfléchissait à une évolution de l'enveloppe, non pas de 3 ou 4 euros, mais de plusieurs centaines de millions d'euros, ce qui remettait complètement en question